La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce soir sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.-

dont ces produits sont réutilisés est criante. Il faut changer de modèle, sortir de la société du jetable. Or ce projet de loi accompagne un système qui ne change pas de modèle ; il installe une politique des petits pas, quand il devrait lancer une course.

Les ménages n'ont produit que 9 % de l'ensemble des déchets français : c'est donc le système entier qui est à revoir, notamment en ce qui concerne les grosses entreprises. Ce projet de loi encourage le recyclage, quand il devrait, au contraire, faire sortir le système du tout-recyclable encourager les produits de seconde main et la réparation- en un mot : nous apprendre à mieux consommer et à mieux réemployer nos déchets. Si l'on veut répondre à l'urgence climatique d'une manière sociale, qui ne laisse personne de côté, il faut apprendre à moins jeter, à réemployer, à réparer et à concevoir des produits durables. L'ordre de priorité

Ces textes européens sont transposés en droit français, mais aucune sanction n'est prévue si les règles de priorité ne sont pas respectées, ce qui laisse une grande liberté dans le traitement des déchets. Cet amendement vise ainsi à créer une sanction lorsque la priorité n'est pas donnée au réemploi. Nous sommes à un moment où

La hiérarchisation des modes de traitement des déchets prévue par la directive européenne du 19 novembre 2008 établit un ordre de priorité : réutilisation, recyclage, valorisation et, en dernier recours, élimination. Transposée à l'article L. du code de l'environnement, cette hiérarchie n'est pas souvent respectée en pratique, alors qu'elle constitue le socle juridique de la gestion des déchets. Des progrès dans sa concrétisation sont constatés auprès des juridictions en cas de contentieux : dans une décision du 28 décembre 2018, rejeté le recours d'industriels contre le décret d'application relatif à la fin de la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux composés de matières biosourcées. Les mesures proposées par les industriels- mise en place de collectes et de recyclages, de programmes de prévention et d'un tri à la source -n'ont pas suffi à remplacer la mesure d'interdiction. Le présent amendement vise donc à instaurer une sanction en cas de non-respect de la hiérarchie.

La réglementation européenne transposée en droit français prévoit que le traitement des déchets doit respecter une hiérarchie privilégiant la prévention des déchets, puis leur réutilisation, leur recyclage et leur élimination. Ce principe général s'applique à tous les acteurs de la gestion des déchets. déchets. Il produit des effets en droit, puisque le juge administratif a pu s'appuyer sur cette hiérarchie dans ses décisions, par exemple pour valider l'interdiction de la commercialisation de certains produits plastiques à usage unique, qui répond à l'objectif de prévention de la production de déchets, alors que les acteurs mettaient en avant l'existence de dispositifs de collecte et de recyclage de ces déchets. Pour autant, il ne paraît pas pertinent de prévoir un régime de sanctions pour l'application de cette hiérarchie,

réutilisation, valorisation, recyclage et, en tout dernier lieu, quand il n'y a pas d'autre solution, élimination. Cette hiérarchie, nous avons voulu la mettre au coeur du projet de loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Je partage donc la volonté qui s'est exprimée qu'on aille le plus loin possible dans le respect de cette hiérarchie.

les caractéristiques environnementales des produits proposés et harmoniser les mentions employées. En effet, l'information des consommateurs peut s'avérer trompeuse, soit par un acte délibéré, soit par négligence ou omission, soit encore parce que les mentions manquent de précision sur le caractère durable, écologique ou naturel des produits ou sur leur réparabilité, leur compostabilité, leur recyclabilité ou leur dangerosité. Il est donc nécessaire d'arrêter ces modalités d'information.

réparer ou recycler tel produit et non tel autre est de toute première importance, et cela facilitera grandement le passage du modèle linéaire actuel- j'extrais, je consomme, je jette -au modèle circulaire- je consomme mieux, je répare, je recycle. L'économie circulaire est un modèle pour la société de demain, avec une création de valeur ajoutée et une baisse de l'empreinte écologique. Elle est une réponse à la crise des déchets, à la nécessité de les gérer, à la raréfaction des ressources. Mais si elle a nombre de vertus,

La communication d'informations telles que l'incorporation de matières recyclées, la recyclabilité des produits et la présence de substances dangereuses me paraît particulièrement utile, de même que l'indice de réparabilité défini à l'article 2 et la simplification des signalétiques de tri prévue à l'article 3. Pour autant, il nous faut nous interroger sur le bien-fondé environnemental de telles mesures. En effet, qui peut sérieusement imaginer que le consommateur, pour chacun de ses achats, contrôlera de lui-même la respectabilité environnementale du produit Si l'objectif est réellement de changer de modèle, il aurait été préférable d'imposer aux metteurs sur le marché des pourcentages d'incorporation de matières réemployables ou recyclables. Permettez-moi également de vous dire que, si l'on peut partager l'intention du Gouvernement en matière de généralisation du logo Triman pour les produits concernés par une filière de responsabilité élargie du producteur, cette mesure signalétique ne réglera pas la question,

Un amendement a été adopté en commission pour prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du produit, de façon globale. De fait, si une information claire sur les déchets engendrés par tel ou tel produit ou telle ou telle commande publique doit être fournie,

de réemploi que nous encourageons tous, il est nécessaire d'identifier la traçabilité de certains matériaux ou matières réemployés ou réutilisés. Je pense- vous n'en serez pas étonnés -au recyclage des pneus, dont certains éléments sont utilisés pour la construction de terrains synthétiques de sport ou de surfaces de jeu pour les enfants, sans que nous ayons d'informations précises sur leur provenance. Les élus locaux s'en inquiètent.

ailleurs, en ce qui concerne les informations sur les substances dangereuses contenues dans tel ou tel produit, il conviendrait de mettre l'accent sur le risque associé à une substance dans certaines conditions

a pour but de faire progresser l'économie circulaire,, notamment, la responsabilité élargie du producteur- nouvelles familles de produits concernés, évolution des modalités de calcul de l'éco-contribution et hausse des flux financiers attendus. Un an après la mise en place de la feuille de route pour l'économie circulaire, ce texte se décline en quatre orientations principales : stopper le gaspillage pour préserver nos ressources, mobiliser les industriels pour transformer nos modes de production, informer pour mieux consommer et améliorer la collecte des déchets pour lutter contre les dépôts sauvages et réduire l'impact environnemental des plastiques. Par ailleurs, il s'inscrit dans le contexte d'une forte demande de la population de replacer l'écologie au centre des politiques publiques, afin de répondre aux enjeux de transition écologique et de respecter les accords de Paris. Pourtant, il semble que, derrière une stratégie de communication bien rodée, ce projet de loi ne soit pas à la hauteur de l'urgence climatique. En effet, les plus grandes avancées environnementales et sociales- bonus-malus écologique, don des invendus, baisse des prix de la réparation -sont formulées au conditionnel, et leur mise en oeuvre est reportée à des négociations ultérieures. De la même manière, on peut regretter que le moratoire demandé par les défenseurs du climat et les « gilets jaunes » pour obtenir la mise en conformité du secteur de la distribution textile et électronique avec l'accord de Paris, ainsi que la limitation de l'expansion illimitée des zones commerciales et d'acteurs de la vente en ligne, comme Amazon, qui augmentent la surproduction le dumping et livrent leurs marchandises par avion, n'aient pas été suivis d'effet. Pourtant, le Haut Conseil pour le climat et les scientifiques avaient solennellement demandé au Gouvernement de revoir à la hausse son ambition, en prenant des mesures pour réduire l'empreinte carbone liée aux importations.

nous nous souvenons de l'amiante : alors, le principe de précaution ne s'impose-t-il pas ? Recycler une matière si problématique a-t-il un sens ? S'agissant d'économie circulaire et de recyclabilité, peut-on continuer sur cette ligne-là ?

! Il y a une multitude d'emballages différents, constitués de plastiques différents qui ne sont pas recyclés et ne le seront pas, parce que l'opération est trop compliquée : cela pose le problème de cette fameuse économie circulaire, qui semble être une illusion. Notre seule planche de salut,

produit. Il nous paraît nécessaire que les consommateurs aient un accès direct à ces informations en magasin, sans être obligés de passer par des plateformes électroniques ou des applications de smartphones.

comme le prévoyait le texte initial. à rendre possible la dématérialisation de l'information à destination du consommateur. L'objectif était bien évidemment de rendre cette information la plus adéquate possible en fonction du produit concerné, afin que le dispositif soit plus flexible. La dématérialisation est essentielle dans un contexte général de réduction des emballages papier et plastique. C'est pourquoi il nous a paru important de sécuriser et de renforcer le dispositif, car il est clair que cette dématérialisation doit être la plus profitable pour le consommateur. Même si l'utilisation d'applications sur téléphone va croissant, comme vient de le souligner notre collègue Joël Bigot, un grand nombre de personnes ne les utilisent pas, et ceux qui les utilisent n'y ont pas recours systématiquement. Gardons donc une souplesse, sans perdre de vue l'objectif premier de l'article : informer le consommateur de manière simple et directe.

par tout autre procédé approprié », qui autorise la dématérialisation de l'affichage des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mis en vente, n'incitera pas les producteurs et importateurs à faire le choix exclusif de ce mode d'information, au détriment du

Toutefois, les informations caractérisant la nature et la gestion de fin de vie des produits, notamment en matière environnementale, sont d'intérêt général : elles ne doivent pas devenir captives d'un intérêt privé ni d'acteurs qui en feraient une source lucrative.

Il serait contre-productif de limiter la portée de l'information à destination du consommateur en réduisant son accessibilité. Évitons donc de privilégier une mise à disposition de l'information par dématérialisation, au détriment d'une communication active.

Cette transparence est nécessaire et voulue par les consommateurs ; elle est attendue dans une relation de confiance, car la défiance est forte et les plateformes accessibles sur smartphone comme les applications fleurissent, ce qui n'est pas ce que nous voulons. Les metteurs sur le marché devraient le comprendre, d'autant que c'est aussi dans leur

produit. S'il est indispensable d'informer les consommateurs sur les ressources utilisées pour fabriquer un produit, sur la nature de l'emballage et sur la réparabilité, des données essentielles manquent sur son impact environnemental, notamment le bilan carbone de son transport et la pollution qu'a engendrée sa production.

conformité avec la philosophie de cet article et pour offrir la meilleure information au consommateur, nous proposons de préciser la proportion du coût de revient de l'emballage dans le prix de vente du produit. En effet, en plus de leur bilan environnemental catastrophique, les emballages coûtent cher et nuisent au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Pour des objets à usage unique, qui finiront nécessairement en déchets, on peut aisément parler d'argent jeté à la poubelle. Une telle mesure permettrait à tout un chacun de réaliser que notre modèle de consommation, reposant sur le jetable, notamment le plastique jetable, avec des suremballages, à un coût financier presque aussi important que son empreinte écologique et représente un gaspillage considérable.

en promouvant un modèle où l'ensemble du cycle de vie des produits est intégré, avec pour objectif de tendre vers 100 % de plastiques recyclés d'ici à 2025. L'intérêt des sacs biodégradables et compostables conformes aux normes en vigueur pour la collecte séparée des biodéchets a été reconnu. Aussi la valorisation organique des emballages biosourcés compostables est-elle une solution qui peut parfaitement s'intégrer aux côtés du recyclage et du réemploi. Toutefois, l'un des freins à la valorisation de ces emballages réside principalement dans la difficulté pour le consommateur de les identifier. Le terme générique de « bioplastique », qui recouvre des réalités très diverses, induit trop souvent le consommateur en erreur. C'est pourquoi il convient de caractériser la fin de vie de l'emballage, en indiquant de manière lisible s'il est compostable ou recyclable. Tel est l'objet du présent amendement.

aux producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets l'information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits. Il tend ainsi à introduire une modification rédactionnelle visant à assurer la cohérence avec la réglementation européenne, qui utilise la notion de « substances

Cet amendement vise à réintroduire les éco-modulations dans la liste des caractéristiques environnementales devant être affichées pour le consommateur. Cette précision a été supprimée en commission sur l'initiative de Mme la rapporteure pour avis, au motif notamment qu'elle serait trop contraignante contraignante pour les producteurs et stigmatisante pour les produits se voyant appliquer un malus. Or ces éco-modulations sont le reflet des efforts consentis par les producteurs pour rendre, comme le précise le nouvel article L. 541-10-3, leurs produits performants d'un point de vue environnemental. En somme, cette information permettra aux consommateurs de mesurer si le produit qu'ils achètent s'intègre ou non dans une démarche vertueuse. Supprimer cette information qui nous semble importante permettra aux producteurs de pouvoir s'acquitter d'un éventuel malus sur leur éco-contribution sans avoir à s'en justifier auprès des consommateurs. C'est un recul évident, tant en matière d'information des consommateurs que du développement d'une économie circulaire ambitieuse.

d'information créé par l'article 1 aux publicités en faveur des produits. L'objectif est double : assurer une information plus complète des consommateurs, qui verront l'information non plus seulement sur les emballages, mais également sur les publicités, et, partant, créer une incitation bien plus forte pour les producteurs à améliorer les qualités environnementales de leurs produits. L'amendement Cet amendement vise à préciser que les modalités d'information des consommateurs sur les qualités environnementales des produits prévues à l'article 1 devront faire l'objet d'une harmonisation au niveau national. L'objectif est de veiller à la bonne lisibilité et compréhension par le consommateur de cette information. En effet, et comme c'est le cas pour l'ensemble des signalétiques d'une manière générale, laisser les producteurs ou metteurs sur le marché totalement libres des modalités d'une telle information en multipliera les déclinaisons, rendant ainsi le dispositif illisible. Il nous semble au contraire indispensable d'en prévoir une harmonisation, dans l'esprit de l'article 3 de ce projet de loi relatif au logo Triman.

Il s'agit bien d'un article-cadre, dont la mise en oeuvre appellera des travaux techniques complémentaires avec les parties prenantes. L'objectif est, en outre, de disposer d'une base légale permettant de lutter contre les allégations environnementales infondées, dont les services de la répression des fraudes

pourra tout à fait encadrer le recours à la dématérialisation en fonction des caractéristiques environnementales concernées ou des canaux de distribution. L'avis est donc défavorable

L'amendement n° 677 vise à remplacer les notions de « qualités et caractéristiques environnementales » par celle d'« empreinte environnementale ». Il nous semble satisfait par un ajout fait en commission visant à privilégier une analyse de qualité environnementale sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Au-delà, nous jugeons préférable de cibler des qualités précises, sans quoi nous risquons d'élargir excessivement le périmètre du dispositif. L'avis est donc défavorable. L'amendement n° 102 vise à imposer aux producteurs de distinguer le coût de l'emballage du coût total du produit. En réalité, les producteurs n'ont pas à communiquer aux consommateurs le coût de revient de leurs produits. Cela reviendrait à afficher la marge qu'ils réalisent au vu et au su de tous,

La compostabilité est une information intéressante, bien qu'assez précise pour être mise au niveau de la loi, étant entendu que l'énumération de qualités et caractéristiques environnementales à l'article 1 n'est pas exhaustive. Néanmoins, un nombre croissant de Français étant intéressés par les pratiques de compostage, il nous paraît intéressant d'ajouter ce point en rappelant que le pouvoir réglementaire précisera les modalités d'application de ce dispositif aux catégories de produits pertinents. Pour cette raison, l'avis est favorable L'amendement n° 333 rectifié vise à informer le consommateur de la présence de plusieurs emballages. Nous partageons pleinement l'objectif de lutte contre le suremballage et avons d'ailleurs proposé en commission d'agir des pénalités financières en fonction du poids des emballages mis sur le marché. Cela nous semble plus utile pour agir sur la production de déchets que de prévoir une information sans doute assez complexe à présenter sur la présence de plusieurs emballages. L'avis est donc défavorable. En commission, sur l'initiative de notre collègue Anne-Catherine Loisier, nous avons précisé que la liste des substances dangereuses serait définie par décret après avis de l'Anses. Il s'agit d'une solution de compromis qui permet tout à la fois de rassurer les producteurs et de répondre aux questions de santé-environnement à l'origine de préoccupations importantes de la part des pouvoirs publics et de la société civile. Cibler exclusivement les substances préoccupantes au sens de la réglementation Reach ferait obstacle à la mise en oeuvre d'autres dispositifs, y compris lorsqu'ils sont prévus par le droit européen, ainsi qu'à des initiatives nationales sur certaines questions sanitaires.

devant obligatoirement être communiquées par les producteurs aux consommateurs, sur l'initiative de notre collègue Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques. De la même façon que la contribution financière de base, ces informations d'ordre technique relèvent du financement de la filière REP et ne constituent pas en soi une information complète ni même lisible sur les caractéristiques environnementales du produit. L'avis est donc défavorable

l'amendement n° 334 rectifié, nous ne voyons pas clairement comment le dispositif d'information sur les qualités et caractéristiques environnementales pourrait s'insérer de façon claire et lisible dans les messages publicitaires sur les produits visés. En outre, il nous paraît utile de rappeler qu'il faut bien distinguer la publicité et les informations données lors de l'achat. La publicité n'a pas à réintégrer l'ensemble des informations, parfois précontractuelles, qu'un vendeur doit communiquer au consommateur lors de sa décision effective d'achat. L'avis est donc défavorable.

est l'avis du Gouvernement ? C'est seulement après la phase d'expérimentation que sera élaboré un décret. Dans la rédaction actuelle, le recours au décret pour définir les modalités d'application permet déjà une mise en oeuvre progressive par modifications successives, après des expérimentations le cas échéant. Cette rédaction permet aussi de démarrer très vite pour les filières qui sont déjà prêtes. C'est pour cette raison que je souhaite en rester à la rédaction actuelle. L'avis est donc défavorable sur l'amendement

C'est effectivement très important, mais la notion d'empreinte environnementale n'est pas la seule information que nous souhaitons révéler au consommateur. Il faut qu'il y en ait plus, et que ce soit plus large encore. Nous voulons, par exemple, pouvoir informer le

Les publicités sont encadrées par des dispositions réclamant leur sincérité, mais elles ne sont pas en général normées. L'article 1 établit un dispositif visant à informer l'acheteur sur le lieu de vente, mais il n'est pas adapté à l'encadrement de la publicité.

tous les amendements procèdent d'une bonne intention, mais parfois le mieux est l'ennemi du bien.

interrogée sur la notion de réparabilité et me suis dit que l'on était en train de faire exactement ce que nos concitoyens nous reprochent, c'est-à-dire que l'on crée un indice qui ne correspond à rien du tout.

Dans la plupart des cas, les consommateurs ne sont en effet pas compétents pour réparer un produit selon les règles de l'art, qui permettent de garantir son bon fonctionnement. Il y va de leur sécurité en cas de mauvaise réparation, mais aussi de la responsabilité du professionnel qui ne sera pourtant pas intervenu sur le bien.

vise seulement à donner une information simple sur la réparabilité du produit. Il n'a pas pour objet d'inciter à la réparation ou à l'autoréparation, mais ne l'empêche pas non plus.

aux vendeurs de leurs produits leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir ». L'alinéa 3 prévoit la transmission d'une partie de ces informations au consommateur, mais ne précise pas que celle-ci doit se faire sans frais. Aussi,

par tout autre procédé approprié ». Ce souci de souplesse se justifie par la nécessaire adaptation aux cas particuliers, selon le type de produit, son type de conditionnement, son lieu de commercialisation. Cela rejoint l'argumentaire que j'ai déjà développé.

! À mon avis, l'obligation faite au vendeur de mettre à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité d'un produit se révèle excessivement contraignante et alourdit inutilement la charge des professionnels de toutes tailles, avec un nombre important d'informations à transmettre au consommateur.

À l'instar de l'amendement n° 332 rectifié que nous avons défendu précédemment, il s'agit de ne pas réserver ce type d'information aux détenteurs de smartphones ou aux publics plus avertis qui pourront, en amont de leur achat, consulter ce type d'information sur internet. Si nous souhaitons renforcer les informations transmises aux consommateurs et les rassurer dans leur acte d'achat, notamment en recourant à des biens durables, ce type d'information doit être consultable directement et rapidement.

ayant permis de l'établir. Cet ajout nous semble important pour tout consommateur qui souhaiterait approfondir cette question avant d'effectuer un achat. À défaut, celui-ci n'aurait accès qu'à une notation sur dix, qui ne lui permettrait pas de bien appréhender les différents enjeux en termes de réparabilité documentation technique, disponibilité des pièces détachées, bref un certain nombre d'informations qui pourraient être importantes pour lui. En vue de modérer la charge pour le vendeur, la commission a bien précisé que cette mise à disposition se ferait

Nous partageons l'objectif de cet article, qui reprend la mesure n° 10 de la feuille de route pour l'économie circulaire, dans la droite ligne des évolutions européennes. encore une fois les modalités concrètes d'application de cette mesure, qui sont renvoyées à un décret pris en Conseil d'État, que nous déplorons. Nous regrettons que le dispositif en reste à de simples obligations en termes d'information.

de produits électroniques ou électriques qui ne disposeraient pas d'un indice de réparabilité satisfaisant. Nous considérons que, pour lutter de manière efficace contre l'obsolescence programmée, il ne suffit pas d'informer le consommateur. Il faut cesser de mettre sur le marché des produits trop peu pérennes et dont la durée de vie est limitée. Les consommateurs, même éclairés, et aux revenus modestes, peuvent porter leur choix sur des produits moins chers, mais moins durables. Nous souhaitons donc créer une véritable exigence de réparabilité auprès des producteurs. Tel est le sens de cet amendement. Quel est l'avis de la commission Il n'est pas opportun d'interdire la mise sur le marché d'un produit au motif qu'il présente un indice de réparabilité trop faible. D'une part, cette mesure serait en contradiction avec une série de normes européennes et constitutionnelles ; d'autre part, l'indice est un dispositif d'information : à charge pour les consommateurs bien informés de consommer en connaissance de cause.

fondement. Nous pouvons néanmoins faire un certain nombre de choses. Je souhaite pour ma part m'appuyer sur les filières REP, sur les éco-organismes, pour développer et structurer l'offre de réparation. Voilà l'enjeu

dans le calcul de la modulation de l'éco-contribution. Les éco-organismes et les producteurs vont s'organiser pour soutenir des réseaux de réparateurs de façon ciblée et

La question de l'omniprésence de la publicité dans notre vie quotidienne est centrale. Cet amendement vise à rendre obligatoire un affichage systématique, qui sensibilise à l'impact de la surconsommation sur l'environnement, sur les publicités faisant la promotion des produits neufs. Il n'est nullement question de culpabiliser le consommateur ou de le rendre seul responsable de cette surconsommation. Celui-ci n'a d'ailleurs généralement pas conscience de l'impact environnemental de sa consommation de produits neufs. Il s'agit non seulement de le responsabiliser, mais également de responsabiliser les publicitaires. Une prise de conscience collective est nécessaire. Nous devons promouvoir un changement culturel pour une consommation plus durable. Quel est l'avis de

Si nous partageons l'idée que la publicité a une responsabilité importante en matière de changement des modes de consommation, cette proposition nécessite que l'on réalise des travaux complémentaires. En visant les publicités en faveur de produits neufs, l'amendement cible en effet un périmètre extrêmement large. La commission y est donc défavorable.

exact que nos concitoyens ne sont pas suffisamment informés des impacts environnementaux de nos modes de consommation. Il est donc important de leur communiquer les bonnes informations qui permettront de lutter contre la surconsommation. C'est tout l'objet de ce projet de loi, et c'est indispensable ! Aujourd'hui,

toute l'importance d'agir sur tous les vecteurs, en amont et en aval, et donc sur la publicité. Si celle-ci peut être réduite grâce à l'allongement de la durée de vie des produits, je crains qu'une telle mesure se heurte à de grandes difficultés dans sa mise en oeuvre pratique.

L'absence d'informations techniques suffisantes et systématiques sur la réparation et l'entretien des biens pour les professionnels est un frein à leur activité.

Les informations techniques relatives à la réparation et à l'entretien des biens doivent être rendues plus accessibles sur le modèle de l'obligation qui existe au niveau européen pour le marché de la réparation automobile. Cet amendement tend à obliger les constructeurs à rendre accessible toute information nécessaire à l'entretien et à la réparation des biens. Cet amendement vise à ajouter aux informations précontractuelles relatives à tous les biens des éléments sur leur entretien et les modalités de leur réparation. En réalité, ces informations relèvent plutôt de celles qui doivent accompagner les biens après leur achat. En outre, l'information préalable à l'achat sera déjà améliorée l'indice de réparabilité prévu à l'article 2. Créer une obligation générale à la charge du vendeur consistant à apporter une information précontractuelle sur l'entretien et la réparation d'un produit nous semble excessif. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable La liste des informations que le vendeur a l'obligation de fournir à l'acheteur étant harmonisée au niveau communautaire, elle ne peut être modifiée par un État membre.

Cet amendement revient sur une disposition que nous avons introduite en commission, sur l'initiative de nombreux groupes, et qui consiste à exclure les emballages en verre du dispositif de signalétique généralisée, au motif des contraintes techniques sur les emballages, d'une part, et d'un geste de tri déjà très bien ancré

de non-traitement, etc. -, une filière qui s'adapte rapidement, mais pour laquelle chaque semaine parlementaire apporte des nouveautés. Cette semaine, c'est le logo Triman

doit être accompagné d'informations sur la nature du geste de tri. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, le verre est le matériau connaissant le meilleur taux de récupération et de recyclage en France : 86,5 % en 2018, selon Citeo.

par tous les pays européens, et une confusion est possible avec le « point vert », lui-même obligatoire pour certaines destinations d'exportation. Pour les mêmes raisons, le Parlement avait déjà exclu les emballages en verre de l'obligation d'imposition du logo Triman lors des discussions sur la loi du 20 décembre de la vie des entreprises. Imposer cette nouvelle contrainte aux entreprises viticoles me semble donc inutile et disproportionné par rapport à l'objectif annoncé d'informer le consommateur que le produit fait l'objet de règles

de l'examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises et motivée par le fait qu'il existait déjà, depuis de nombreuses années, un système de collecte et de recyclage du verre atteignant, cela a été souligné par ma collègue Nathalie Delattre, des taux exceptionnels, tout en étant bien identifié par les consommateurs. Avec la rédaction proposée, le dispositif s'appliquerait notamment aux entreprises productrices de vins et spiritueux utilisatrices de verre, qui informent déjà largement les consommateurs.

La plus-value de l'apposition du logo Triman sur les emballages ménagers en verre étant limitée, l'introduction de cette contrainte n'apparaît pas efficiente au regard de l'objectif visé. la prolifération des déchets par une meilleure information des consommateurs sur la gestion du tri doit être encouragée, mais il nous incombe de veiller à ne pas adopter des dispositions superfétatoires. relève d'une consigne de tri définie par un décret du 23 décembre 2014, excluant les emballages ménagers en verre de son champ. Mes chers collègues,

comment avez-vous fait pour vous mettre aussi rapidement à dos cette filière- une filière importante ? Par des prises de décision

L'article 3 vise à généraliser le logo Triman afin d'améliorer l'information délivrée aux consommateurs sur les règles de tri. Si cet objectif est plus que louable, il nous semble important de renforcer également la transmission d'une information sur les possibilités de réemploi et de réutilisation du produit. Ainsi, le consommateur pourra guider son achat en toute connaissance de cause quant au devenir éventuel dudit produit au moment où il souhaiterait s'en défaire. Nous pourrons de la sorte encourager des comportements d'achat plus vertueux, en incitant les consommateurs à s'orienter vers des produits réparables ou réutilisables, en d'autres termes vers des produits plus durables. le présent amendement, nous proposons donc que les informations accompagnant la signalétique sur les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit fassent état des possibilités de réemploi ou de réutilisation.

à prévoir que tout produit générateur de déchets mis sur le marché à destination des ménages fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet d'un réemploi ou est susceptible de le faire. Cette signalétique permettra de sensibiliser davantage le public sur le réemploi. Nous espérons qu'elle permettra de mieux guider les consommateurs vers un acte d'achat plus vertueux et éco-responsable.

de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément.

Ces quatre amendements, rectifiés à la demande de la commission, tendent à compléter utilement l'information sur le geste de tri, en prévoyant que, en cas de produits comprenant plusieurs éléments relevant de modalités de tri différentes, ces modalités seront détaillées pour chaque élément. L'avis est donc favorable. Quel est l'avis du Gouvernement

souvent d'harmoniser et de simplifier toutes ces règles. Mais, pour certains produits, il peut être pertinent de prévoir une alternative à la mention de cette indication sur le produit lui-même ou sur son emballage.

La signalétique obligatoire incluant les modalités de tri sur le produit, l'emballage ou la notice est un dispositif contraignant, allant à l'encontre de l'objectif de simplification de la vie des entreprises. À titre d'exemple, elle poserait des difficultés techniques importantes à l'ensemble des secteurs du jouet et de la puériculture. de la marque Playmobil. En effet, en raison de la complexité et de la diversité des produits et de leur emballage, il faudrait prévoir des blocs messages systématiques et différents pour chaque référence, sur un marché qui en propose, chaque année, plus de 50 000 nouvelles. La nouvelle signalétique pourrait en outre nuire à la lisibilité des avertissements de sécurité, déjà trop nombreux sur les emballages, cela a été rappelé à plusieurs reprises par mes collègues. Dans de nombreux cas, il faudrait agrandir les emballages, voire ajouter des notices en papier, ce qui serait contre-productif au regard de l'objectif visé de réduction à la source des déchets. La mise en oeuvre de la signalétique commune obligatoire sur le produit, son emballage ou la notice induirait des coûts importants pour les industries françaises du jouet et de la puériculture. Pour ces motifs, il est essentiel de maintenir la possibilité de dématérialisation de cette signalétique. La parole

pour les entreprises exportatrices produisant en France, en l'absence d'un système de tri harmonisé au sein de l'Union européenne. Il importe que les règles soient communes afin de ne pas contraindre à de coûteux changements d'étiquetage en fonction du pays de destination. Par ailleurs, l'apposition obligatoire de la signalétique de tri renvoie à des contraintes techniques pour des entreprises mettant sur le marché des produits de petite taille, vendus sans emballage ou notice ou avec un emballage réduit au maximum et saturé. Dans de nombreux cas, il faudra ainsi créer ou augmenter la taille des emballages, voire ajouter des notices en papier en vue

qui, ne l'oublions pas, a pour finalité d'améliorer les gestes de tri et, donc, la qualité de la collecte séparée sur de nombreux produits. J'ai bien entendu vos arguments relatifs à la place qu'occuperait un logo supplémentaire sur nos produits,

La signalétique proposée à l'article 3 devrait être accompagnée d'informations précisant les modalités de tri. Or la loi relative à la transition énergétique prévoit l'harmonisation des consignes de tri. Il convient donc d'attendre que cette dernière soit effective avant de créer une nouvelle obligation d'étiquetage. C'est pourquoi cet amendement tend à renvoyer l'entrée en vigueur de cette disposition à une date fixée par décret.

et électroniques et pour les biens d'ameublement. Là encore, nous ne pouvons que souscrire à l'objectif, visant tant à orienter le choix de consommation vers des produits plus durables qu'à favoriser le geste de réparer plutôt que de racheter du neuf. Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face. La réparabilité, en l'état actuel des modes de production et d'achat, n'est pas toujours chose aisée. Tous les équipements ne sont pas réparables à l'infini, et nous savons, notamment dans le secteur de l'électroménager, qu'il n'est pas rare de voir des pièces détachées coûtant plus cher que l'achat ou le rachat d'un produit neuf. Par ailleurs, il existe aussi un risque non négligeable de devoir importer des pièces détachées dont l'empreinte carbone peut être interrogée. Dans ce cas, l'objectif environnemental visé s'en trouverait fort amoindri.

le marché des pièces visibles automobiles. Il a été décidé, en particulier, d'abaisser de vingt-cinq à dix ans le délai de protection pendant lequel certaines pièces automobiles restent sous monopole des constructeurs. Cela participait de la lutte contre la vie chère outre-mer et contre l'abus de position dominante exercée par des oligopoles. a entraîné, pendant des années, la multiplication du phénomène des véhicules hors d'usage- les fameux VHU -devenu un véritable fléau aux Antilles, en particulier en Martinique. Imaginez donc, 60 000 véhicules- 20 000 en Martinique ; jusqu'à 30 000 en Guyane -présents sur la voie publique ou sur des propriétés privées et s'apparentant à des épaves. Ces chiffres sont considérables. Aucune commune de la Martinique n'est épargnée par les VHU, même s'il est vrai que le nombre d'épaves de voiture est plus important dans le centre de l'île. Le décret du 28 avril 2017 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage, couplé à l'arrêté du 28 avril 2017 définissant le contenu et les modalités de mise en oeuvre du plan d'actions des producteurs automobiles en application du 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement, tend à résorber le problème et prévenir une éventuelle reconstitution du phénomène. Ainsi, 3 117 VHU collectés depuis le mois d'avril 2018 ont été enlevés, puis éliminés en Martinique. Il y a une amélioration, mais cela reste insuffisant.

nous y reviendrons en temps voulu. Ainsi, l'amélioration de l'information du consommateur quant à la disponibilité des pièces détachées et du recours à des pièces issues de l'économie circulaire en cas de réparation

l'amendement n° 232 rectifié. Cet amendement tend à apporter plusieurs modifications pour augmenter la réparabilité des produits, améliorer l'information transmise aux vendeurs et aux consommateurs, ainsi que la protection de ces derniers, et clarifier les obligations des fabricants ou importateurs. Premièrement, il tend à fixer une obligation de fournir des pièces détachées pendant une période de dix ans après la fin de la mise en disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. Deuxièmement, il vise à prévoir que le fabricant ou l'importateur informe le vendeur professionnel de la non-disponibilité temporaire et exceptionnelle et précise la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées sont indisponibles.

des amendements précédents, cet amendement vise à imposer au fabricant ou à l'importateur de fournir les pièces détachées pendant une période de dix ans à partir de la fin de la disponibilité des biens sur le marché, autrement dit la fin de la commercialisation du produit par le fabricant lui-même.

de connaître sans ambiguïté l'échéance de fin des engagements de durée de disponibilité des pièces détachées dont un produit bénéficie.

allant jusqu'à l'inscription dans les documents commerciaux, bénéficient de la connaissance exacte de tous les éléments qui composent l'engagement de durée du metteur sur le marché. Le

à la disponibilité des pièces détachées, afin de mieux orienter les choix des consommateurs vers les équipements électriques et électroniques durables parce que réparables. Avec cet amendement, nous proposons d'aller plus loin dans cette direction. L'obligation d'information sur la disponibilité des pièces détachées

l'article L.111-4 du code de la consommation n'oblige pas les fabricants ou importateurs à informer les vendeurs que les pièces détachées ne sont pas disponibles, ce qui induit une mauvaise information du consommateur. Nous proposons donc de clarifier la rédaction du présent article en indiquant que, lorsque l'information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées sont réputées indisponibles, comme le prévoit le texte, et que cette information est affichée comme telle au consommateur afin d'éviter toute confusion. Nous espérons que cet amendement, que nous pourrions qualifier de clarification ou de simple précision rédactionnelle, sera adopté. Ces dispositions vont dans le sens d'une meilleure information du consommateur et donc d'un essor, comme nous pouvons l'espérer, du secteur de la réparation des pièces électriques et électroniques, notamment par un renforcement du recours à l'économie sociale et solidaire.

du consommateur quant à la disponibilité de pièces détachées avant l'achat d'un bien. Pour l'heure, cette information est rendue obligatoire par la loi dans le seul cas où le fabricant aurait transmis l'information au distributeur.

Ces dispositions s'inscrivent dans la continuité d'un amendement adopté en commission afin de favoriser la réparation du matériel médical en ayant recours à des pièces issues de l'économie sociale et solidaire.

Les amendements identiques n 232 rectifié, 548 rectifié et 657 tendent à imposer une période de disponibilité de dix ans pour les pièces détachées nécessaires à l'utilisation de l'ensemble des équipements électriques et électroniques et des équipements d'ameublement. L'article du code de la consommation modifié par l'article 4 vise à informer le consommateur quant à la disponibilité des pièces détachées et, le cas échéant, la période de disponibilité. Il s'agit de permettre au consommateur de décider d'acheter tel ou tel bien en tenant compte des enjeux de réparation, de réparation, et non d'imposer au fabricant ou à l'importateur une période de disponibilité des pièces ; ce laps de temps varie non seulement selon les catégories de produits, mais aussi entre chaque produit. Il revient ainsi à l'acheteur de faire son choix en tenant compte, notamment, de ce critère.

: nous ignorons le délai moyen de disponibilité sur les différents marchés concernés et, en conséquence, la faisabilité d'une telle évolution. N'oublions pas non plus qu'il s'agit, dans plusieurs cas, de marchés européens, voire internationaux. de ces amendements ne précise pas quelle serait la conséquence en cas de non-disponibilité des pièces détachées sur une telle durée, situation probable pour une part non négligeable De manière générale, sauf pratique qui pourrait paraître abusive ou trompeuse, ma philosophie est d'améliorer l'information du consommateur pour qu'il puisse disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à un achat éclairé sur l'impact environnemental du produit. Mais je suis soucieuse de ne pas imposer aux entreprises

l'amendement n° 309 peut créer une contrainte pour les fabricants, mais elle permettra également d'améliorer le recours à la réparation, en fournissant des informations plus précises aux vendeurs et aux réparateurs professionnels, ce qui nous semble aller dans le bon sens. Nous émettons donc un avis favorable.

La commission n'a pas examiné ce sous-amendement ; mais à titre personnel j'y suis favorable, dès lors qu'il tend à maintenir l'apport principal de l'amendement de notre collègue, consistant à demander au fabricant de transmettre au vendeur le détail des pièces de rechange disponibles.

loi. La rédaction consolidée de cet article indique : « Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indisponibles à l'utilisation des biens sont réputées non disponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l'achat du bien. Il n'y a pas d'ambiguïté quant à l'obligation créée par ce texte, à la charge du vendeur, d'informer expressément le consommateur de la non-disponibilité des pièces, y compris lorsqu'elle sera déduite de l'absence d'éléments transmis par le fabricant aux vendeurs.

tend à préciser qu'en l'absence d'éléments transmis par le fabricant sur la disponibilité des pièces détachées le vendeur communique par tout moyen au consommateur la mention « aucune assurance sur la disponibilité des pièces détachées ». Sauf exception, il ne revient pas à la loi de préciser les formulations ; c'est au pouvoir réglementaire de prévoir, le cas échéant, une distinction d'affichage entre l'absence d'éléments sur l'indisponibilité et l'indisponibilité avérée. En outre, la modification que nous avons adoptée en commission sur l'initiative de notre collègue Joël Bigot, afin de clarifier l'obligation pour le fabricant d'informer le vendeur quant à la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces, devrait résorber cette difficulté.

coïncidera dès lors avec le délai imparti au distributeur pour réparer un produit dans le cadre de la garantie légale de conformité. Nous avons opté pour cette solution de compromis équilibrée en concertation avec la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, Mme Loisier. Nous émettons, en L'amendement n° 344 rectifié vise à imposer une disponibilité de dix ans pour les pièces détachées nécessaires à l'utilisation des équipements médicaux.

concerne les informations que le fabricant doit fournir au vendeur : il est utile de laisser au fabricant le choix d'indiquer au vendeur la période de disponibilité des pièces ou alors

d'empêcher un producteur, un importateur ou un vendeur d'équipements électroniques de réserver à un réseau de réparateurs agréés la fourniture

posent des obstacles pratiques à une réparation rapide, efficace et économique des produits pour inciter les consommateurs à racheter plutôt qu'à réparer.

nous partageons l'objectif de non-discrimination des réparateurs par les fabricants, mais, à nos yeux, le droit en vigueur comporte déjà des dispositions générales faisant obstacle aux discriminations dans les relations entre fabricants et réparateurs. Dès lors, cet amendement est déjà satisfait, et j'en demande le retrait. Quel est

L'option d'utilisation de pièces détachées telle que prévue par ce projet de loi impliquerait que les circuits de distribution mettent à disposition toutes les pièces de rechange demandées par le consommateur.

est à M. Joël Bigot. L'article 4 prévoit que tout réparateur d'équipements électriques et électroniques doit permettre au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire en lieu et place des pièces neuves. Nous faisons nôtre cet objectif, qui s'inscrit dans la continuité de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, Toutefois, nous proposons de préciser cette rédaction en indiquant que le réparateur ne devra pas seulement permettre, mais encourager le recours à de telles pièces. Il s'agit d'une nécessité dans la logique d'une économie circulaire efficace où tous les acteurs de la chaîne, du producteur au consommateur en passant par les intermédiaires, comme les réparateurs, orientent notre système vers davantage de réemploi et moins de consumérisme. L'article 4 impose aux réparateurs de cinq catégories d'équipements électroniques de proposer à leurs clients d'utiliser des pièces de rechange issues de l'économie circulaire. Le contenu de cette obligation, notamment les catégories de pièces concernées, sera déterminé par un décret en Conseil d'État.

détachées dans le secteur de l'automobile : très logiquement, le réparateur n'est pas tenu de proposer des pièces de rechange issues de l'économie circulaire si elles ne sont pas disponibles.

L'article 4 crée une obligation de moyens, et non de résultat. En l'absence de filière de disponibilité de pièces, le réparateur sera dispensé de cette obligation. L'inquiétude de notre collègue n'a donc pas lieu d'être, et il nous semble préférable de favoriser l'économie circulaire. L'expérience dans le secteur automobile montre qu'un tel dispositif facilite la structuration du secteur du réemploi et les partenariats avec les filières de réparation. Cher collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. Quel est

Cette disposition étant inscrite à l'article 13, le présent amendement n'est donc pas bien placé. Sur le fond, en anticipant une adoption de la loi au début de 2020, il nous semble indispensable de donner un délai suffisant aux réparateurs

? Monsieur le sénateur, je partage tout à fait votre ambition d'aller vite pour améliorer l'information du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées et sur la possibilité d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire.

Cet amendement, issu d'une concertation avec le collectif Halte à l'obsolescence programmée, a pour objet de renforcer la portée, et donc l'effectivité, de l'indice de réparabilité. Comme le souligne le Livre blanc intitulé « 50 mesures pour une consommation et une production durables », depuis le 1 mars 2015, les distributeurs et les fabricants sont tenus d'afficher la durée pendant laquelle ils s'engagent à fournir les pièces détachées des biens qu'ils commercialisent. commercialisent. Toutefois, plus de 60 % des vendeurs n'informent pas correctement sur la disponibilité des pièces détachées. La

et la durée de disponibilité de chacune d'entre elles et de prévoir la possibilité de sanctions pour pratique commerciale trompeuse en cas de fausse déclaration.

commission ? Le projet de loi prévoit déjà un régime de sanctions administratives en cas de manquements à ces obligations d'information. Il ne nous semble pas souhaitable de faire dès à présent référence à un régime pénal et à une qualification de ces manquements comme délits sanctionnés d'une peine d'emprisonnement, en particulier pour une obligation nouvelle

du Gouvernement ? Il faut sanctionner les pratiques commerciales trompeuses des fabricants ou des vendeurs qui mentent aux consommateurs sur l'indice de réparabilité et la disponibilité des pièces détachées. Il est absolument intolérable qu'il puisse

confiance. Tout ce qui abîme la confiance doit donc être combattu ! Toutefois, la rédaction actuelle de l'article L.121-2 du code de la consommation vise déjà des pratiques commerciales trompeuses qui portent sur les caractéristiques des produits, et plus particulièrement sur leurs qualités substantielles.

et surtout l'environnement, du fait des quantités importantes de déchets ainsi générées. La garantie légale de conformité est un outil au service de l'allongement de la durée de vie des produits. Pour inciter les producteurs à mettre sur le marché des produits plus durables et pour protéger les consommateurs de pratiques visant à réduire la durée de vie des produits, l'amendement vise à allonger à dix ans la garantie légale de conformité, qui est aujourd'hui de deux ans. Ainsi, les consommateurs constatant qu'un produit est impropre à l'usage attendu, y compris plusieurs années après l'achat, pourront bénéficier de cette garantie.

Les dépenses des Français consacrées aux biens de consommation ont été multipliées par trois depuis 1960. Cette évolution est due, entre autres causes, au système de l'obsolescence programmée. Nous parlons bien de système, car il a été démontré que les produits étaient conçus pour durer le temps de la garantie.

Une étude de l'UFC-Que Choisir indique que, dans l'hypothèse d'un allongement de la garantie de deux à cinq ans, testé sur trois produits électroménagers- lave-linge, four, réfrigérateur -, celui-ci entraînerait une augmentation du prix du bien comprise entre 1 % et 2,9 L'étude conclut que cette hausse mesurée serait vraisemblablement couverte, pour le consommateur, par les gains économiques liés à la diminution du renouvellement et à la gratuité de la réparation. Une étude de l'Institut de l'industrie et des systèmes dingénierie conclut pour sa part que « de meilleures conditions de garantie ont pour résultat accroissement des ventes ». Enfin, selon le rapport Libaert, l'instauration d'une garantie de cinq ans ne pénalisera pas les entreprises françaises, car la mesure s'appliquerait à l'ensemble des produits vendus en France, quel que soit le fabricant. L'argument d'une possible distorsion de concurrence envers des distributeurs français qui verraient échapper une partie de leur clientèle, celle-ci préférant s'approvisionner à l'extérieur de nos frontières, n'est

Ces amendements visent à porter la durée de la garantie légale de conformité de deux à cinq ans ou de deux à dix ans en vue de l'allongement de vie des produits. Il s'agit de propositions discutées depuis plusieurs années, puisqu'elles avaient été évoquées dès la conférence environnementale de 2013. pour la transition énergétique, en 2015, le Parlement avait demandé au Gouvernement un rapport sur l'opportunité d'une telle extension. Remis en avril 2017, ce rapport recommande de porter ce sujet au niveau européen, dès lors que la durée de la garantie légale de conformité fait l'objet d'une harmonisation à deux ans dans la directive « consommation » de 1999. Il est possible pour les États membres d'aller au-delà, mais, eu égard à l'existence d'un marché européen intégré, il est peu probable qu'une initiative nationale isolée conduise à une évolution significative de la conception des produits. La marge d'ajustement risque alors d'être le prix de vente. En outre, la commission attire l'attention de l'ensemble des auteurs des amendements sur le fait qu'il s'agit d'une évolution extrêmement structurante, pour ne pas dire bouleversante, pour l'ensemble de notre industrie. Nous sommes donc très réservés sur le principe d'une telle modification sur la base d'une initiative nationale isolée, d'autant que la plus-value apportée par une telle extension fait encore l'objet de débat. La position de la commission sera la même sur l'ensemble des amendements visant à allonger la durée de la garantie légale de conformité : avis défavorable aux amendements n 506 rectifié,